La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème l'État territorial entre Mirages et réalités de membres de la délégation aux collectivités territoriales. Je vous rappelle que dans ce débat. Le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire. De prendre la parole immédiatement après je à chaque orateur pour une durée de deux minutes. L'orateur disposera alors à son tour du droit d'répartis pour une minute. Madame la Ministre, vous pourrez donc si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé sa place dans l'hémicycle. La parole et tout d'abord à l'orateur de la délégation qui a demandé ce débat. Madame, Françoise Gatel, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Le titre du débat qui nous réunit ici cet après-midi peut paraître provocateur l'État territorial entre mirage et réalité. Mais cette apparente provocation est en fait. Forte de sa vérité puisque. Il rend compte des incertitudes de graves qui pèsent sur le rôle de l'organisation de l'État dans nos territoires, question qui a été mise en évidence pendant la crise sanitaire, le malaise est vraiment palpable tant auprès des élus locaux mais ça ça n'est pas une surprise au 1er rang duquel des mères mais aussi des usagers et aussi ce malaise s'étend aux agents de l'État eux-mêmes pourtant l'État déconcentrer a fait l'objet de multiples attentions depuis une quinzaine d'années. C'est même l'un des principaux champs de réforme de l'action publique. Les acronymes n'ont pas manqué pour désigner des politiques qui ont touché les services déconcentrés de l'État. Je les cite pour mémoire, la rehab la Real pardon la MAP. La PPNG cette cascade de de réformes me semble traduire des tâtonnements et des coups de volant un peu brusque, à l'exemple du, du préfet, le préfet de département, Pierre angulaire de l'État déconcentrer. Il a vu ses marges de manoeuvre réduite par l'éruption si je puis dire du préfet de région puis ses compétences réaffirmer avec toutefois toujours un pouvoir d'évocation et donc de reprise du sujet par le préfet de région et voici désormais que le préfet sera fonctionne Alizée fondu dans un corps plus large que celui de la préfectorale, qui vient de disparaître. Alors cette succession saccadé de réforme est le signe, je pense qu'on est d'accord là-dessus tous d'un défaut de vision et d'une faiblesse dans l'évaluation de ces politiques successives. Vous savez, madame la Ministre, l'évaluation des politiques publiques est au coeur de la culture du Sénat singulièrement de sa délégation aux collectivités territoriales pour ce que ce qui les concerne, mais aussi de la commission des lois, aucune des réformes que je viens d'égrener n'a fait l'objet d'une évaluation ex Post digne de ce nom. Tout s'est passé comme si les idées préconçues les remèdes miraculeuse miraculeux pardon et les intuitions plus ou moins judicieuse prenait le pas sur la rigueur et l'objectivité tirant ce constat d'un déficit d'évaluation la délégation aux collectivités territoriales s'est particulièrement investi sur le sujet et je veux saluer l'excellent travail de nos deux collègues. Agnès Canayer Éric Kerrouche qui ont conduit ces derniers mois une mission d'information remarquable extrêmement fouillé et rigoureuse. Leur mission a conduit à un rapport intitulé A la recherche de l'État dans les territoires parce que c'est un peu Indiana Jones. Quand on est élu local et ça n'est pas un énième rapport un marronnier, on va dire dans un domaine qui en compte beaucoup mais bel et bien une boussole pour l'avenir avec une vision très claire de ce que doit être l'État dans nos territoires et tout autant de ce qu'il ne doit pas être nos 2 collègues n'ont pas hésité à prendre directement le pouls du corps préfectoral, au travers d'un sondage et il n'est pas si fréquent. Madame la Ministre que les préfets sous-préfets se livre ainsi à coeur ouvert si je puis dire sur leur vécu professionnel et je veux d'ailleurs remercier au nom de la délégation. Monsieur le ministre Darmanin, qui a rendu possible cet exercice de consultation des préfets sous-préfets inédit mais fructueux. Et d'ailleurs. Pouvez-vous rappeler quand vous allez rentrer au ministère de l'Intérieur monsieur Darmanin que nous serons très heureux de lui remettre en mains propres. Ce rapport cette consultation des membres du corps préfectoral, s'est accompagnée d'un sondage auprès des élus locaux. Alors cette seconde consultation. Révèle on va dire un intérêt extrêmement important, mais encore plus fort quand on rapproche le résultat des 2 études car il se trouve que le point de vue des élus locaux et des membres de la préfectorale se rejoignent sur de nombreux points, ce qui ne manque pas de rendre ce rapport fort pertinent. La comparaison des points de vue fait ressortir plusieurs points saillants. Un accord sur le fait qu'une réforme territoriale de l'État et souhaitable. Par ailleurs, ce sont les représentants de l'État qui dénonce le plus le rythme de la réforme. 85% d'entre eux contre 64% des élus locaux. Et si le sentiment d'une absence d'associations réforme est très forte chez les élus, plus de 80%. Il est loin d'être négligeable chez les représentants de l'État puisque 43% d'entre eux estiment que. Il y a un manque d'associations de consultation des préfets à ces réformes, enfin et c'est très révélateur. Seul un représentant de l'État sur 4 estiment que la réforme de l'organisation territoriale de l'État est efficace. Est-ce pour autant à dire qu'un grand soir de l'État, territorial est attendu pour reprendre les termes de nos collègues qui en parleront sûrement Canayer et Kerrouche. Nul besoin d'un nouveau Big-bang territorial. Au sein de l'État, territorial en revanche l'État a besoin de retrouver son efficacité dans le dernier kilomètre et jusqu'à l'ultime citoyen pour y parvenir, nous sommes convaincus ici au Sénat, renforcé par l'analyse de la crise sanitaire de la pertinence d'un échelon de l'État au niveau départemental, il nous semble que pour grand nombre de défis. C'est un bon niveau mais pour bien vivre ce qu'on a appelé le couple mère préfets de département. Celui-ci doit pouvoir compter sur un accompagnement de l'État qui change sa culture en disposant de plus de moyens. C'est un état qui accompagnent qui facilite et qui permet et non pas un État tatillon contrôleur voire parfois avec certains services qui interprète à sa manière erronée par par me pardonnez-moi de le dire l'esprit du législateur. Les rapporteurs parleront de leurs suggestions de leurs questions, mais moi je voudrais souligner une suggestion révolutionnaire qui fait un peu le buz dans le milieu. Il s'agit pour moi d'une proposition extrêmement pertinentes puisque c'est le rattachement des préfets au 1er ministre il n'y a pas d'autre moyen d'avoir une cohésion des politiques de l'État et de leur application et madame la mini-si la République est une et indivisible. Il me semble que l'État doit l'être tout autant et que l'État parle d'une seule voix et que le préfet soit un chef d'orchestre de me semble une idée pleine de bon sens. Madame la mini-je suis sûr que nous avons par ce rapport. De quoi susciter une intense réflexion. Je rappelle que notre débat s'inscrit dans un calendrier qui est marqué par la volonté du président du Sénat d'avancer à l'attention du gouvernement de nouvelles propositions en matière d'efficience de l'action publique, notamment par le biais de la décentralisation et la déconcentration. À l'issue d'un travail qui associe l'ensemble des groupes politiques du Sénat nos échanges vont alimenter cette ambition et je ne doute pas que nos échanges Madame la Ministre vont aussi alimenter la réflexion du président de la République car je me suis laissé dire que le président de la République que penser qu'il était urgent d'adapter l'architecture. Institutionnelle pour plus d'efficience. Nous ne cessons de réformer de corriger sous des espèces de lifting ou de pansement avec tout cela, nous souffrons d'un mal extrêmement profond qui consiste par ses réformes successives. On va dire à. Les élus locaux empêcher l'action publique dont nos concitoyens et besoin et surtout toutes les réformes territoriales que nous avons travaillé ont carrément éludé la question existentielle c'est, quid de l'État. Quelles sont les fonctions de l'État. Quels sont ses ses compétences et je cesse madame, je n'ai de cesse Madame la Ministre de rappeler que nous devrions mettre fin à ses aventures hasardeuses de recomposition parce que nous partageons tous ensemble et je n'en doute pas un seul objectif c'est l'efficience de l'action publique dans une relation de confiance entre l'État et les collectivités. Merci madame la présidente. Et avant de de passer aux différents orateurs, je vais demander à Madame la mini-si elle souhaite. Intervenir pour le moment non parce que vous avez la possibilité de le faire si vous le souhaitez, après chaque orateur ou oratrice.

Madame la Ministre, madame la présidente. Mes chers collègues. Un État n'existe que sur un territoire donné, avec une population et une organisation institutionnelle durable. L'État et donc par naturel territoriale l'expression État territoriale et donc tout tout il était, il existe un lien indéfectible entre l'État et les services déconcentrés et ses services déconcentrés. D'une part et les collectivités territoriales d'autre part. L'expression État territorial traduit la difficulté à concevoir l'État à l'échelle locale qui deviennent plus une variable manières managériales d'un État soucieux de faire des économies qu'une perspective de développement territorial penser sur le temps long. Les nombreuses réformes engagées lors des 20 dernières années illustrent les difficultés à répondre aux 2 questions majeures sur le rôle de l'État. quelles doivent être les rapports entre l'état et les élus locaux, premièrement et deuxièmement quelle est l'organisation optimale de l'État à l'échelle locale. Je rappellerai d'abord une évidence qui tend parfois à être oublié l'administration territoriale de la République est assuré par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'État. D'après la loi de 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Si l'État est unitaire sur l'organisation territoriale passe par une des concentrations effective au service des collectivités territoriales et de la population. La réforme continue des services de l'État et les principales réformes comme l'a rappelé la présidente. Adopté emporté sur la révision et la modernisation de l'action publique avec par exemple la RGPP les lois MAPTAM et notre dans l'objectif d'améliorer la situation, mais sans vraiment y parvenir, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir un État locales moins dispersé et recentré sur ses missions en ce sens la proximité et l'accessibilité de l'État doivent être renforcées dans le cadre départemental en concertation avec les élus locaux. Deuxièmement, le nombre de réformes crée des difficultés d'assimilation pour y pallier, je pense nécessaire de renforcer le rôle de l'État de mieux associer les élus locaux aux réformes des services déconcentrés. Je pense également que le rôle du préfet de département est primordial dans la mise en oeuvre des réformes et la la stratégie du dernier kilomètre afin que les décisions soient prises au plus près des citoyens dans une logique de subsidiarité permettant d'envisager la différenciation territoriale. Sans nier le rôle du préfet de région. Le préfet de département doit être une ressource pour les élus locaux, notamment des petites communes, un coordinateur et un pilote des pilotes des politiques Pivot entre l'État national et local, le préfet de département doit pouvoir disposer des ressources humaines et budgétaires suffisantes, ce qui n'est pas malheureusement pas plus toujours le cas depuis plusieurs années au contraire de cette tendance. Je partage l'idée qu'il faut réarmer until intelligemment. D'abord, avec plus de moyens humains. Une demande qui émane du corps préfectoral corroborée par le dernier des chiffres édifiants, en adaptant l'organisation des services déconcentrés certains services sous tutelle ministérielle comme les Dreal ou OFB dispose d'une autonomie excessive leur pouvoir de décision pose des problèmes concrets dans la mise en oeuvre des politiques publiques par exemple sous les, les énergies renouvelables sous la protection contre les risque de prédation et. Ses services déconcentrés devrait pour des raisons que j'ai déjà évoqué être sous l'autorité du préfet. Au total le démembrement ou l'éclatement de l'État un opérateur et autres agences ne conduit plus à la simplification territoriale qui est paradoxalement le maître mot des réformes depuis 15 ans enfin les services déconcentrés doivent conserver au niveau de compétence pour l'exercice de leur mission d'ingénierie territoriale ça m'éteindre je terminerai pour mentionner les risques que font peser la fonctionnarisation. Des préfets l'augmentation du préfet thématiques et le délaissement des sous-, préfectures sur l'organisation territoriale de l'État. Pour que l'État territorial ne soit pas une on est plateforme. Il est donc nécessaire de renforcer les services déconcentrés de l'État en suivant des principes simples qui ont été rappelés proximité compétences sous l'autorité du préfet et dans le cas du département il y a donc nul besoin de unième d'un énième Big bang territorial simplement de revenir aux fondamentaux de l'administration territoriale de l'État. Je vous remercie. Merci. Donc Madame la Ministre vous si vous souhaitez intervenir pour 2 minutes. En réponse à l'orateur. Allez-y, Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Je. Vous remercie pour cette première question qui me permet de rappeler quelques fondamentaux, même si bien sûr, les choses peuvent toujours être améliorés. Alors comme l'indique la constitution le le préfet est le représentant de l'État et de chacun des ministres du gouvernement, c'est lui qui met en avant les politiques de l'État, avec l'ensemble des services qu'ils soient placer ou non. Sous son autorité directe. On a bien vu sa capacité à piloter tous les services durant la crise Covid, où le couple mère préfet a fait preuve de son efficacité au service de nos concitoyens. Vous vous en félicitez. Et nous aussi. Ah, parfait. Donc alors on diverge excusez-moi j'avais compris qu'on était. Sur ce couple mère-préfet tout à fait en phase. Le 2ème, point sur lequel Monsieur le Sénateur. On est parfaitement en phase, c'est sur le fait que l'État est par essence territoriale. Et donc. Comme je viens de vous le dire l'interlocuteur naturel est bien connu des élus. C'est le préfet, c'est le représentant de l'État et de chacun des ministres du gouvernement. Les élus le savent aussi peuvent compter sur son équipe de proximité les sous-préfets d'arrondissement c'est parce qu'il joue un rôle essentiel que l'État a décidé de les renforcer. Pour rappel, cinq sous-préfecture que plus tard dans d'autres réponses je vous laisserez ont rouvert leurs portes et une nouvelle sous-préfecture a été créé en Guyane. 30 postes de sous-préfet ont été créés par redéploiement des postes de sous-préfet à la relance. Dans des départements ruraux et dans ce qui compte une équipe préfectorale peu nombreuses. Donc en renforçant l'État territoriale, le gouvernement fait le choix de renforcer les interlocuteurs naturels des élus. Pour faciliter son action et lui donner de nouvelles marges de manoeuvre. Dans le cadre de la loi 3DS le préfet désormais, délégué territorial de plus d'opérateurs qu'avant l'Ademe l'OFB et en plus de l'ANRU là c'était Elana qui existait déjà. Des mesures de simplification ont aussi été prises en sa faveur. Le préfet de département peut désormais signer des décisions d'attribution de ces deux décident en lieu et place du préfet de région mais. Comme, comme vous aurez la possibilité mais c'est normal hein on se règle sur la règle du jeu comme vous aurez la possibilité d'intervenir après chaque orateur, il faut que ces se tenir au deux minutes mais. Non non mais c'est chacun s'. Apprivoise la règle du jeu, c'est normal Monsieur Anglade vous avez la possibilité de vacances donc je vais donner la parole maintenant à notre collègue Colette Mélot pour le groupe les indépendants pour cinq minutes.

Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. La la quête de l'Union, l'unité nationale est ancienne. Déjà à la veille de la révolution française, les Français invités à rapprocher administration de leurs administrés. Les cahiers de doléances ont participé à instaurer une nouvelle organisation territoriale visant notamment à permettre à chacun de pouvoir se rendre au chef-, lieu de son département Anne une journée à cheval. Située à moins de 30 minutes en voiture et non à cheval du domicile de chaque Français les maisons France services se sont multipliés en France. Élément fort de la traduction de l'État, territorial ces espaces couvre même les zones les plus isolées via des solutions mobiles comme par exemple dans les Terres montagneuses de la Corse. C'est une bonne chose car toutes les solutions sont bienvenues pour maintenir une offre de services publics de proximité. Les retours de terrain sont globalement bons, et les Français se les approprient progressivement. Nous en sommes tous convaincus ici la diversité de nos territoires fait la richesse de la France en milieu rural ou urbain en montagne ou à outre-mer les élus locaux n'ont pas les mêmes attentes et leurs habitants n'ont pas les mêmes besoins dans une logique de différenciation les politiques publiques doivent correspondre au mieux aux spécificités de notre territoire, nous devons raisonner à travers une une grille de lecture plurielle. Je souhaiterais également parler de l'accompagnement des élus la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la haine, c'était en 2020. Visite à fluidifier les relations entre l'État et les collectivités territoriales et à faciliter la réalisation de leurs projets locaux. Lors de l'examen du budget pour 2023. Notre groupe salué l'augmentation des dotations qui lui sont destinées. Nous venons d'apprendre que les effectifs humains de la haine c'était vont être augmentées dans les préfectures, cela paraît être une excellente nouvelle qui va dans le bon sens. Un récent rapport sénatorial pointait justement du doigt le manque d'implication de certains préfets selon ce même rapport, l'agence est trop éloignée du terrain et des préoccupations des élus. Elle doit au contraire remplir sa mission d'outil facilitateur. Nous le savons les solutions viennent généralement directement du local, l'État doit t'apporter une oreille attentive aux remontées du terrain et accompagner les élus face aux défis qu'ils surmontent quotidiennement. Madame la Ministre, le Tour de France des régions que vous réaliserez avec les dirigeants de l'Agence devrait participer à poursuivre le dialogue. Nous espérons que les conclusions que vous en tirerez nourriront de manière effective, les politiques publiques conduites par votre ministère. L'État territorial est basée sur 2 piliers les collectivités décentralisées et des administrations déconcentrées. Ce système est amené à évoluer régulièrement pour s'adapter aux évolutions de notre pays et aux besoin des élus. Ces dernières années les réformes territoriales se sont succédé. La dernière en date la loi dite 3DS s'inscrit dans la digne voie de la décentralisation, tout en apportant son lot d'ajustements techniques. Pour s'y retrouver. Les élus doivent avoir accès à des relais d'information facilitateur souples et simples d'accès. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer. Comment l'émission des agents des préfectures et des sous-, préfectures pourraient être amenée à évoluer pour mieux répondre à l'impératif de proximité avec les élus locaux. Par ailleurs, quels dispositifs sont prévues pour prendre davantage en compte l'an la vie des citoyens dans l'organisation des services déconcentrés et dans l'élaboration des politiques publiques à visée territoriale. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice mélo.

La façon avec laquelle on renforce les moyens de l'État en région. Et puis pour finir les maisons France service sur le sujet de la haine. C'était si vous avez lu notre communiqué de presse hier. Nous nous sommes grandement inspiré du rapport du Sénat. Ils nous ont remis. Les les 3 sénateurs. Sont venus nous remettre ce rapport que moi j'ai perçu de façon très positive malgré des quelques critiques que nous avons pris comme des axes d'amélioration et sur lesquels nous sommes appuyés pour décider. À la fois de doubler les effets. Motif de ANC c'était en région et en même temps les mettre dans les sous-, préfectures pour être au plus proche puisque vous appelez de vos voeux une plus grande proximité donc sur le sujet de la haine. C'était, elle a été créée. En janvier 2020 n'a que 3 ans. Il reste comme je vous l'ai dit des axes d'amélioration. sur lesquels nous travaillons ensemble et vous l'avez cité. Nous allons entreprendre avec le président bouillon et directeur général un tour de France des régions parce que vous appelez de vos voeux que je vous dise comment on peut améliorer cette proximité de la haine c'était mais aussi des agents qui sont en préfecture. C'est bien l'objet de ce Tour de France des régions que le président bouillon va entreprendre et qu'avec Christophe Béchu et maman nous allons embarquer pour essayer de voir quelles sont. Les les les leviers sur lesquels on peut agir en matière de proximité. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure pour une plus grande proximité mais je veux quand même rappeler les 2 axes de travail, des moyens de l'État en région. 5 sous-préfecture. Aucun emploi n'a été supprimé sur le périmètre T E en 2021 2022 la création de 350 ETP supplémentaires qui est prévu en 5 ans, dont 43 dès cette année 30 postes de sous-préfet créer par redéploiement des postes de sous-préfet à la relance. Je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le gouvernement renforce son partenariat avec les collectivités. Je peux pas vous redire ce que j'ai dit sur la une, Mais je veux vous dire parce que j'aurai l'occasion de le redévelopper ce partenariat dans d'autres questions qui m'ont été posées, mais je veux conclure en saluant vos propos sur les maisons France service qui effectivement. Sont. d'une vraie efficacité sur notre territoire avec un budget qui a été alloué de 200 maisons de France service supplémentaires dans les territoires pour toujours et encore plus de proximité, merci. Merci, madame la Ministre Madame Mellow une minute. Merci, merci Monsieur le Président Madame la Ministre je vous remercie pour les différents éléments que vous venez de nous donner. Ont tout d'abord. Les améliorations qui avait été apportées sont vraiment vont vraiment dans le bon sens et puis il nous espérons beaucoup que celle que vous nous annoncerez après votre tour de France iront aussi dans le même sens. Merci. Merci la parole est maintenant à notre collègue Thomas Dossus du groupe écologiste solidarité et territoires. Merci monsieur. Le président, madame la présidente de la délégation aux collectivités territoriales Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans un monde idéal, les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État devrait être en mesure de répondent parfaitement aux besoins des habitantes et habitants comme aux besoins des élus de leur territoire. L'action publique serait facilitée par une organisation claire fluide et efficace. De la gouvernance à l'échelon local, les actrices et acteurs publics locaux serait valorisé ils disent. Poserait de compétences et de moyens conséquents pour jouer leur rôle et les services publics serait accessible à toutes et tous, force est de constater que ce doux rêve n'est pas la réalité. Les nombreux échanges que chacun d'entre nous peut avoir avec les élus locaux nous font la démonstration quotidienne du mirage l'État territoriale à proprement parler. L'excellent rapport d'information sur l'état dans les territoires fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales. Et à la décentralisation par mes collègues Agnès Canayer Éric Kerrouche en fait une démonstration limpide. Prenons déjà l'exemple des réformes des collectivités et des services déconcentrés. Les années passent et ces réformes se multiplient au gré des conjonctures politiques la révision générale des politiques publiques, la modernisation de l'action publique et la loi 3DS en sont autant de preuves et venant d'une métropole à statut particulier celle de Lyon. Je peux vous dire que la lisibilité de l'action publique, qu'elle soit étatique ou territoriales reste de plus en plus floue pour nos concitoyens pour. Si le vent des réformes à brouiller la compréhension de l'action publique. S'il y a un point commun à ces réformes, c'est qu'elles ont été construites souvent de façon brouillonne et avec une concertation très limité des premières. Les premiers concernés, c'est-à-dire les élus et assez peu les représentants de l'État déconcentrer. Il faut entendre aussi une forme de fatigue des élus de ces réformes incessantes qui n'ont rien clarifié le rapport d'information de l'État dans le territoire l'explique bien plus de 4 élus sur 5 estime ne pas avoir été suffisamment associés aux différentes réformes. Pour les préfets et les sous-préfets ce chiffre s'élève à 43%. Déjà en 2016 un autre rapport d'information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Précisait que l'association aux réformes des acteurs de terrain demeure insuffisante aux yeux de la majeure partie des élus locaux et des syndicats qui ont été auditionnés. Mais comment mener une réforme efficace des politiques de décentralisation et de déconcentration. Si les autorités locales et les administrations concernées ne sont pas suffisamment concerté. Si l'État reste trop à distance. La réponse c'est qu'on ne peut pas le rapport de mes collègues le démontre comme celui. Tout récent, vous l'avez dit sur la sur la une, c'était le Les réformes ne correspondent pas à leurs attentes et ne résolvent pas un certain nombre de leurs problèmes. Les moyens principalement humains manque parfois dans les territoires et ce manque se fait ressentir sur l'ensemble des politiques publiques en 2011. Les effectifs publics des directions départementales interministérielles s'élevait. À 39.796 agents. Mais ces direction on n'en comptait plus que 25.474 en 2020, soit une chute de 36%. Les préfectures ne sont pas en reste et ont connu une baisse similaire. Ce n'est pas le statut des agents comme on a pu entendre déjà ce matin mais bien l'austérité à bas bruit qui a sclérosé notre capacité à mener des politiques publiques. Gilles et répondant aux besoins. La situation des. Services publics, hôpitaux, écoles et autres guichets administratifs délétère dans de nombreuses régions et en particulier dans les zones rurales. À ce titre, près d'un maire sur 2 de communes de moins de 1000 habitants, estime que l'offre de services publics sur un territoire est défaillante. C'est d'autant plus compliqué pour ces maires des petites communes qui sont souvent isolés et qui ne dispose pas des mêmes ressources que les grandes collectivités. Ces dernières sont mieux représentées au sein des agences comme les ARS ou Lana et elles peuvent mobiliser des réseaux importants, ce qui n'est pas le cas des élus de petites communes. Alors que faire. Si l'État. Est un mirage pourrait-il devenir réalité. Il faut commencer par respecter l'ensemble des parties prenantes et inscrire la concertation, le dialogue au coeur de l'action publique. Le lien de relation de confiance durable et parfois à retisser d'urgence et plus finement, avec l'ensemble des actrices et acteurs du territoire je rejoins les préconisations de mes collègues sur la nécessité d'une concertation nationale avec les élus en amont de toute réforme des services déconcentrés de l'État ou des collectivités territoriales. Avec le groupe écologiste. Nous sommes convaincus que le principe de subsidiarité doit être consacré tout comme la différenciation territoriale, cela ne doit pas cependant être fait, comme l'a proposé le gouvernement au travers de la loi 3DS. Qui en plus d'échouer à clarifier les compétences à accélérer la tendance de l'État se défausser de certaines de ses prérogatives sur les collectivités. Or les collectivités territoriales doivent avoir les moyens d'agir. Il doit y avoir un voyage. Plus enfin dans la répartition des effectifs préfectoraux notamment dans les sous-, préfectures, la proposition qui me semble la plus pertinente et forte du rapport de mes collègues mais elle n'est pas nouvelle, propose de passer enfin d'une logique de contrôle de légalité. Tu es à celle de conseil aux collectivités territoriales. Mais l'État est-il prêt à sortir d'une logique de contraction de ses effectifs pour s'adapter à cette demande notamment au plus près des territoires parfois démunis en matière de relais préfectoraux à l'ingénierie de leur projet. La clé de l'État, territorial se situe à mon sens dans la réponse à cette équation. Je vous remercie. Merci cher collègue. Et pendant que vous. Rejoignez votre place, je vais demander à Madame la Ministre de répondent si elle le souhaite. Pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur de suce. Je vais m'éloigner de des notes que que qu'ils m'ont été préparés parce que. En effet, beaucoup de choses ont déjà été dites dans les réponses aux premières questions L'État territorial Mirage évidemment je ne partage pas ce point de vue. Comme vous le savez je suis. Pendant six mois aller beaucoup sur le terrain en tant que secrétaire d'État à la ruralité. J'ai rencontré environ 40 préfet de département. Et ses préfets de département dire qu'aujourd'hui. Leurs équipes et eux-mêmes sont un mirage. Non seulement même qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le prendrais pas très bien mais en plus je suis allée à la rencontre d'élus locaux dans ces départements environ une soixantaine par département à chacune de mes VO et je me suis jetée dans cette arène en sachant que, oh combien effectivement les élus locaux sont en demande de plus plus plus de proximité, être rassurés et donc cette exigence elle me paraît totalement légitime, j'étais maire jusqu'au 7 juillet mais je peux pas vous dire que c'est un mirage, parce que beaucoup de choses sont déjà fait dans le sens de plus de dialogues et plus de proximité, je pense qu'aujourd'hui le corps préfectoral. Les services de l'État en région en quasi-totalité sont au service des élus locaux et la première phrase si c'est pas la première, c'est la seconde ou la troisième que que les élus me me dise quand je me trouve à dialoguer avec eux, c'est je vais vous dire à quel point le préfet, les services, le sous-préfet est efficace, tous les élus locaux et j'ose vous le dire franchement et s'il y a des endroits dans lequel les services de l'État ne donne pas satisfaction à à à nos élus, j'en suis extrêmement surpris, ça peut toujours arriver de ci de là mais en tout cas, globalement on a l'impression que du service de l'État et et moi qui arrive, moi je suis le gouvernement et et et je suis là pour évidemment parler Dusan parler de choses. Qui sont un peu contraignante, mais les services de l'État sont à leurs côtés, donc pas de Mirage pour moi. Vous appelez de vos voeux, quelque chose qui nous tient corps et sur lequel nous travaillons, c'est la différenciation. Je veux dire à quel point les lois passées comme la loi montagne par exemple où le pouvoir dérogatoire du préfet qui peut déroger, pour s'adapter à une situation sur le terrain, l'organisation de Lyon qui a montré que les spécificités ont fait qu'une organisation spécifique a été mis en place en tout cas le président de la République et le gouvernement sous l'autorité de la Première ministre. Nous voulons plus de différenciation donc on répond favorablement à votre appel et pour finir, vous dire que les réformes, vous dites les réformes les réformes en fait elles se sont arrêtées les réformes donc oui il y en a eu beaucoup par le passé et vous avez raison mais on est en phase de stabilisation et donc que je m'arrête parce que j'ai dépassé, bon. Merci madame la ministre. Monsieur dessus je voulais ajouter un mot. Non. Donc, la parole est maintenant à notre collègue Bernard buis pour le groupe RDPI. Monsieur le président. Madame la ministre, madame la présidente de la délégation. Mes chers collègues. Il me semble qu'en 2023 l'État territoriale en France relève davantage de la réalité que du mirage en effet ces dernières années, nous avons assisté au réarmement de l'État dans les territoires un réarmement concret et financier sur le plan concret comment débattre de l'État, territorial sans évoquer les 2538 Maison France service elle représente à mes yeux le symbole d'une proximité retrouvée dans nos territoires ruraux entre l'État et nos concitoyens. Comme l'a souligné le récent rapport sénatorial de notre collègue Bernard Delcros. L'intérêt du programme France service est désormais indéniable, il réside essentiellement dans la proximité et la dimension humaine de l'accompagnement apporté aux usagers grâce aussi au déploiement de 4000 conseillers numérique à l'heure où le digital. Encore parfois. Une partie de la population de l'accès aux services publics. Force est de constater que le réseau France service est aujourd'hui saluée par une majorité d'usagers et d'élus locaux. Pas moins de 93,4% des usagers sont satisfaits de leur démarche dans ces espaces. Quant aux 520 élus locaux. Interrogé par la plateforme de consultation du Sénat. Seuls 6 5 % considèrent que le dispositif n'est pas pertinent. Même certaines communautés de communes pourtant réticente en 2019 lorsque le réseau fut créée, ont pu voir que les espaces France services répondent aux besoins et aux attentes de la population. Mes chers collègues lors du lancement de l'agenda rural le programme France service était une priorité aujourd'hui. Ces maisons sont une réalité et surtout le programme est un franc succès à l'image de l'espace France service de dans mon département de la Drôme qui enregistre 5581 demandes annuelles, justifiant ainsi la sollicitation. Pour une nouvelle labellisation dans le territoire du Diois, le renforcement de l'État, territorial s'illustre également depuis ces dernières semaines dans certains territoires Nantua dans les rangs ce soir en Haute-Vienne Château-Gontier en Mayenne Clamecy dans la Nièvre Montdidier dans la Somme Saint-Georges de l'Oyapock en bus Guyane fin 2022, nous avons été témoins de la réouverture ou de la création de sous-préfecture en France. Quand je pense au réarmement de l'État, territorial. Je pense également à la création de 200 brigades de gendarmerie prévus dans la Lopmi, programmée en janvier 2024. La cartographie des implantations réalisées en lien avec les préfets et les collectivités sera d'ailleurs publié très prochainement. Je pense enfin à la relocalisation de service de DGFIP dans 50 villes médiane sélectionné depuis 2022 21. Nous avons pu en bénéficier en Drôme et en Ardèche. Salut mon collègue ardéchois. Autant d'exemples concrets qui démontrent, pourquoi l'État territorial n'est plus un mirage mais bel et bien une réalité perceptible et salué mais comme chacune et chacun le sait, dans cet hémicycle le réarmement de l'État, territorial ne peut être complet, que si les financer. C'est d'ailleurs un marronnier dans cet hémicycle. Ainsi, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, le programme administration générale et territoriale de l'État qui porte notamment les moyens du réseau préfectoral des services placés sous l'autorité des préfets de région et des directions départementales interministérielles a connu une hausse de crédit de 13,3% par rapport à 2022. Une hausse qui viendrait renforcer de manière inédite, les moyens et les effectifs de l'administration territoriale de l'État à hauteur de de 79 milliards d'euros. Une évolution note enfin à plus de 20 ans de réduction systématique des effectifs départementaux et nous le souhaitons à la lente érosion des Liens entre l'État et nos concitoyens. Autre motif de satisfaction de ce budget le nombres draps Parentis dans le réseau de l'administration territoriale devrait continuer à croître en 2023. Rappelons que 622 apprentis étaient présents dans ce réseau au 31 décembre 2021. Ils étaient 2 fois moins nombreux en 2020. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons assisté au rejet des crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État par le Sénat. Toujours est-il que l'État territorial dispose aujourd'hui de moyens financiers supplémentaires non négligeables et c'est ce choix budgétaires qui permet le déploiement concret du réarmement sur tous les territoires. Cela étant, il reste encore beaucoup à faire et de nombreux progrès peuvent être réalisés pour renforcer l'État territorial dans notre pays alors que pourrions-nous faire de mieux. Nous avons des marges de manoeuvres en terme d'ingénierie de l'État. L'Agence nationale de la cohésion des territoires doit je crois renforcer ses Liens avec les élus. En réponse à la remise du rapport d'évaluation de notre délégation hier vous avez Madame la Ministre souhaiter un nouveau souffle pour l'ingénierie des collectivités dans l'objectif de faire de la haine. C'était un interlocuteur de proximité et du quotidien pour les élus locaux communs, ce nouveau siffle pourrait-il se concrétiser par ailleurs l'efficacité et bien évidemment au coeur de la perception en matière de service public. Le baromètre de l'action publique a été une formidable création mais dans quelle mesure les citoyens se saisissent de cet outil. Comment pourrions-nous le développer. Vecteur de cohésion sociale. J'envisage enfin d'État territorial comme un État facilitateur travaillant de manière complémentaire avec tous les acteurs locaux au service 1er de nos administrés aussi dans quelle mesure l'État territoriale pourrait-il aller davantage vers les administrés. Autant de réflexion que je souhaitais vous partagez à l'occasion de ce débat et qui rappelle que l'État territorial n'est ni un mirage ni une chimère, c'est bel et bien une réalité dont nous devons renforcer l'existence. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre pour 2 minutes. plusieurs sujets je serai très courte sur le sujet de la haine, c'était que j'ai déjà développée. Je vais être amené encore à développer pour juste zoomer sur ce sujet la haine c'était sur l'ingénierie. C'est un outil d'ingénierie dans les territoires, ça me permet de répondre à Monsieur le sénateur qui est déjà parti. Sur les les petites communes. Nous travaillons à l'heure actuelle pour compléter le dispositif c'était sur un programme qui viserait accompagnées en ingénierie. Les petites communes, il est cité comme étant effectivement des communes qui requérait beaucoup d'attention. Nous y travaillons Hélène c'était va agir auprès de ses petites communes vous avez cité les maisons France service je ne redirai pas comme vous l'avez très bien dit à quel point elles sont utiles à quel point elles descendent dans un niveau de capillarité avec les 2600 francs service dans nos territoires et donc vous redire à quel point il il faut que dans vos territoires vous fassiez savoir que nous avons encore 200 maisons France service disponible si possible des véhicules, parce qu'on s'est aperçu que elle permettait de couvrir un véhicule une dizaine de villages et c'était extrêmement précieux 3ème sujet, vous dites que le renforcement de l'État, territoriale, il passe et le réarmement il passe par des moyens humains. Je les ai largement développé, mais il passe aussi par des. Budgets et ses Budgets ont été votés et vous l'avez rappelé, pour la première fois avec une augmentation de plus de 13% pour finir vous avez pour la première fois évoqué le sujet du baromètre. Je veux dire à quel point le président de la République a souhaité. Mettre en place dès 2021, ce baromètre de l'action publique qui porte en son sein des objectifs et de l'évaluation que vous appelez tous de vos voeux et qui sont. Pour nous extrêmement important ce baromètre présente aux Français pour chaque politique des indicateurs chiffrés précis décliné pour les 101 départements. De métropole et d'outre-mer et portant sur la situation initiale en 2017 ou la date de lancement sur la réforme. Le niveau d'avancement à date et l'objectif que nous poursuivons. À l'époque donc pour 2022 depuis sa mise en ligne il a reçu ce baromètre 2 12 millions de visites avec en moyenne 90.000 visites par mois pour vous dire à quel point il est utile. Vous appelez, vous appelez de vos voeux que nous le pérennisons. La réponse est oui, monsieur le sénateur, nous le période. Relisons et nous le rend malade sont aller tendant à 60 politiques prioritaires du gouvernement. Merci. Merci madame la ministre. La parole est maintenant à notre collègue. Ah pardon. Monsieur Buy voulait ajoutant. Oui juste 2 mots pour vous remercier Madame la Ministre par rapport aux précisions que vous apportez, autant sur le baromètre que sur le développement de la haine. C'était sur mon petit territoire merci. Merci. Merci. Donc maintenant, la parole est à dans le trop collègue Thierry Cozic du groupe socialiste, écologiste. Ces républicains. Pour quatre minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, au travers de la loi dite la terre, on retrouve le lien de l'État, territorial entre l'État et ses services déconcentrés. Et les collectivités territoriales mais comment définir cet État territoriale. Nous pourrions évoquer les services rendus par l'État au travers de ses missions et les services publics ainsi que les services au public. Les réformes de l'État, territorial résulte d'une sédimentation de phases successives de la décentralisation. Les réformes se sont enchaînés ces dernières années en dépit d'une intention louable résidant dans la volonté d'améliorer le fonctionnement des services pour répondre au mieux à la demande de d'État dans les territoires. Force est de constater que le compte n'y est pas. Et le résultat est perfectible, notamment au regard de la baisse des moyens de l'État dans les territoires trop souvent prélude d'une dégradation à bas bruit de l'offre de service public. Le tout couplé à l'extrême difficulté pour les élus locaux à identifier le bon a-t-il interlocuteurs dans les méandres de l'administration territoriale. Les conséquences de ces réformes systématiquement dépourvue d'évaluation ont ainsi fini par jeter le trouble, tant chez les élus locaux que chez les chez les agents de l'État eux-mêmes. Nous avons perdu le lien entre les élus et les services déconcentrés de l'État qui ne s'y retrouve plus. À la défaveur de la crise Covid. Le couple mère préfet a été remis en lumière mais il n'est pas superfétatoire de s'interroger sur son efficacité. Tous 2 représentants de l'État est dotée de la compétence générale ils incarnent la République dans les territoires. Le maire et le préfet coproduisent l'action publique au quotidien. Le préfet est le représentant du gouvernement. De l'État et du territoire qu'il administre céderont dont le savant dosage entre ces 3 fonctions qu'il doit être jugé. De fait, une étroite collaboration entre élus et préfet nécessaire mais à quel prix. Les communes gèrent de plus en plus de compétences pour lesquelles elles n'ont pas de moyens affectés. Malheureusement ces charges nouvelles sont loin d'être compensée par un État qui pourtant délègue de plus en plus ses pouvoirs. Mais continue à vouloir les contrôler à distance. la poursuite du processus d'érosion de la fiscalité locale est à l'oeuvre. Par le biais de la suppression de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation. Le tout couplé à la baisse des impôts de production, les collectivités semblent frappés par une recentralisation rampante de leurs ressources. Symbole des relations orageuses entre le président Macron et les maires. La suppression de la taxe d'habitation a été vécue comme injuste et inique pour la plupart de nos élus locaux. Je rappelle que cette suppression aura eu pour effet de faire passer de 54% à 35%. L'autonomie des intercommunalités. Cette réforme ne trahissez que trop bien la vision du candidat Macron qui n'a jamais caché son peu d'intérêt pour l'autonomie fiscale qu'il considère comme un combat d'arrière-garde au regard de plusieurs exemples européens ou l'absence de fiscalité propre n'empêche pas les collectivités d'être puissante. Je le crois sincèrement. Il n'y a pas de pouvoir politique sans pouvoir fiscal. Avec les réformes mises en oeuvre ces dernières années. Le gouvernement considère les collectivités territoriales comme des sous-traitants de l'État. J'en veux pour preuve le systématique basculement sur des dotations dont une partie est indexé sur le produit d'impôts nationaux. De fait, nos collectivités sont placés à la merci du gouvernement qui peut modifier comme bon lui semble. Les dotations et compensations en loi de finances. Soyons honnêtes dans cette affaire. En réalité c'est la pensée dominante de Bercy qui l'a emporté cette vieille idée tenace qui anime la haute administration française. Considérant souvent que l'autonomie fiscale locale n'est pas souhaitable, car les élus locaux ne saurait pas gérer les finances publiques. Alors Madame la Ministre comment penser un État territoriale qui n'est pas un mirage. On peut parler d'État territoriale sans lui octroyer les leviers financiers autonome lui permettant d'administrer ce même territoire. Sans changement de doctrine de la part du gouvernement. Pensez-vous Madame la Ministre que l'idée d'État territorial est encore un sens Girondins. Merci cher collègue. Et pendant que vous reprenez votre place je cède la parole à la ministre pour 2 minutes. Merci monsieur le président. Monsieur mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Cozic. Vous abordez le le le le sujet de l'autonomie. Des collectivités. Je vais évidemment. Pas partager votre analyse de la situation. Je pense au contraire qu'il faut tordre le cou à l'idée d'une perte d'autonomie financière des collectivités. et laissez-moi finir a augmenté en 20 ans. Ainsi le taux d'autonomie financière a augmenté de 10 pour le bloc communal. Entre 2003 et 2020, il est passé de 59% à 75% pour les départements et de 41,6% à 73,9% pour les régions. C'est pas le lieu pour le développer mais je me tiens très sincèrement monsieur le sénateur, à votre disposition pour approfondir ce sujet et partager nos analyses. Ensuite il y a eu des suppressions d'impôts, il faut s'en réjouir. Le gouvernement l'assume la suppression de la taxe d'habitation, c'est plus de pouvoir d'achat pour les Français et les Françaises, la suppression de la CVAE. C'est plus de compétitivité pour nos entreprises. Oui ce sont des marqueurs de notre gouvernement et je ne peux pas partager votre sentiment quand vous dites le peu d'intérêt que le président Macron. Qu'on. Accorde à l'autonomie des collectivités locales. Je vous dis non, par contre je vous. Souligne à quel point il a un très fort intérêt, le président Macron pour la suppression des impôts. Alors effectivement la compensation, hé bien le le sujet qui nous préoccupe tous les élus locaux nous pensons que la préservation de l'autonomie des collectivités que vous remettez en cause, de par la suppression de ses impôts et je comprends parfaitement votre analyse. Elle nous pensons qu'elle a été prise en compte dans la compensation des suppressions d'impôts locaux car les recettes fiscales perdues ont été remplacés par d'autres recettes fiscales du même montant et de même nature. Je me, je vous propose pour ne pas être trop longue de. Approfondir ce sujet un peu technique avec vous à votre convenance. Merci.

Même les données, il faut qu'on les croise, on a, on n'a pas les mêmes. N'a pas les mêmes résultats après sur la suppression de la taxe d'habitation. Certes il y a une volonté du gouvernement de vouloir supprimer les impôts donner du pouvoir d'achat. Sauf que, pourquoi pas si si vous le souhaitez après faudra gérer aussi comment. Nos, nos enfants, nos nos petits-enfants auront à gérer le stock de dettes aujourd'hui qui est une première qui une première chose. Comment le finance. deuxième en plus j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, cette réforme elle est plutôt dirigée en faveur d'une classe très Trezeget plutôt qu'en faveur de des gens qui ont qui ont un peu moins de moyens. Et dernier aspect. Supprimer le lien entre le citoyen et la commune. Je pense que c'était une erreur. Merci cher collègue. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue Michelle Gréaume pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, n'a cessé de travailler d'auditionner des acteurs et des associations pour trouver des réponses, des solutions à ces réflexions qui ne date pas d'aujourd'hui, celle de la place de l'État, territorial de sa présence et de son action au sein de notre République. Cet État territoriale qu'il est encore trop absent encore trop observateurs encore trop à l'écart des réalités de nos collectivités et des demandes de nos habitants, madame la Ministre, l'État doit s'appuyer sur ses services déconcentrés en leur donnant les moyens d'agir, c'est uniquement de cette manière-là que l'administration territoriale de la République pour assurer sa mission de service public auprès de celles et ceux qui en ont besoin au quotidien. À coups de réformes successives. Vous avez éloigner l'état de nos territoires de nos collectivités territoriales, ça fait plus de 10 ans que l'État se désengage à coups de fermeture préfectorale. De baisses budgétaires qui ont des conséquences drastiques sur la gestion quotidienne au sein des services déconcentrés de l'État. Alors oui, la réalité celle-ci l'égalité républicaine promise par l'État est une illusion a mirage. Pourquoi un désengagement si fort de l'État. Se sont comme trop souvent les collectivités territoriales qui subissent état de réformes souvent sans les ressources et l'j'nourri nécessaire. Il y a quelques mois encore nous étions interpellé par les maires de nos départements. Concernant les demandes de passeports et de cartes d'identité nationale. Les administrations ne disposait pas de moyens humains et financiers pour assurer ce service public. Sans compter les délais de traitement lancer en préfecture pour les mêmes raisons. Je ne vous parle même pas de celles et ceux qui ont besoin de renouveler leur titre de séjour pour continuer de travailler pour obtenir un emploi pour se loger dignement. Les files d'attente, dès 6h du matin dans les préfectures n'en finissent pas, voilà la réalité de l'État, territorial. J'aimerais m'arrêter mais la réalité nous rattrape. Alors pour compenser le manque de moyens, on privilégie la déshumanisation avec la forte dématérialisation qui impacte le service public. Prenons l'exemple des maisons France service qui ont été créés pour accompagner cette dématérialisation mais qui sont confrontés à des obstacles les Liens sont rompus avec l'administration, les agents n'ont pas la formation adéquate et de ce fait ne peuvent garantir un service public à la hauteur pour les usagers. Amer sur deux de communes de moins de 1000 habitants, estime que l'offre de service public sur son territoire est défaillante. La crise sanitaire à témoigner de l'importance et de la nécessité d'associer les élus locaux dans les décisions qui impacte les collectivités territoriales. De ce fait le lien avec les représentants de l'État, les préfets et plus que jamais nécessaire. La place du préfet du département de sous-préfecture est importante. Le couple mère préfet doit vraiment exister aujourd'hui 4 élus locaux sur 5 estime ne pas avoir été suffisamment associés aux différentes réformes des services déconcentrés de l'État, l'État doit mettre à disposition une ingénierie efficace et efficiente afin d'accompagner les élus locaux, au quotidien, notamment lors de la construction de grands projets. Durant les discussions autour du projet de loi de finances, nous avons défendu cette volonté de transparence, notamment dans l'attribution de subventions de l'État avec la DETR, et la. Il faut rendre visibles les critères instauré des commissions qui permettent d'expliquer. Chaque projet et motiver les refus pour bénéficier du fonds vers les élus locaux vont devoir compter sur le préfet pour qu'ils juge c'est le projet s'inscrit dans une démarche écologique ou non. Encore une fois un travail en amont d'échange de concertation entre les élus locaux et le préfet s'euros ah dispensable donc Madame la Ministre les politiques et réformes imposées par l'eau ne permettront à l'État, territorial d'exister et de jouer le rôle qu'on lui demande, celui d'assurer une mission de service public auprès de nos habitants habitants et de nos territoires. Il faut que le préfet soit identifié et il faut qu'il soit à l'écoute de celles et ceux qui occupent le terrain au quotidien. Il faut que les moyens alloués soit à la hauteur des besoins. Il faut de l'horizontalité dans la pratique, pour que nos territoires soit réellement réarmer comme le souhaitait l'ancien ministre monsieur comment comptez-vous renouer ce lien rompu entre l'État et ses territoires prendrez-vous en considération les réflexions menées au sein de notre délégation merci. Si. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Vous utilisez des termes forts désengagement déshumanisation. Bien sûr je ne les partage pas et j'espère que ce n'est qu'une perception et que. Notre sentiment, les actions que nous conduisons font que. Ce désengagement cette déshumanisation n'est pas réalité. je vais citer quelques éléments que et et et vous donner quelques éclairages complémentaires à ce que j'ai déjà donné mais les maisons France service accompagné des conseillers numériques. C'est tout sauf de la dé-humanisation. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de ces 50 dernières années, même dans l'histoire de notre République 2600 lieu dans lequel dans lequel nous délivrons 9 service d'état dans lequel accompagnés par un conseiller numérique et tout ça financé entre 50% et 2 tiers par l'État mis dans les collectivités territoriales pour aller au plus près du citoyen pour donner des renseignements sur, je vous dis neuf service d'état ensuite sur le service et vous avez raison. Aux étrangers. L'État soutient, et depuis déjà plusieurs mois un effort continu pour réarmer les services étrangers, le nombre d'agents qui sont affectés, a augmenté de 63 pour 112 ans pour répondre à l'urgence et favoriser un service à l'usager de qualité mais vous le savez comme moi les, le contexte de, de crises géopolitiques et migratoires au cours de ces dernières années, entraîner une augmentation significative de la charge qui pèse sur les services étrangers et notamment en matière de séjour et d'asile, donc ça pourrait être mieux et et vous entendez dans tous mes propos qu'on on pourrait toujours faire mieux mais en attendant, je suis là pour vous rappeler ce qui est déjà fait et le travail remarquable, je veux le saluer, qui est fait par nos préfectures nos préfets et nos sous-préfet nos secrétaires généraux de préfecture en région parallèlement la dématérialisation sur ces démarches étranger au travers de. L'association nationale des étrangers en France devrait permettre à terme d'alléger la charge des services étrangers de gagner en efficacité et en services vis à vis de ces étrangers. Je vous remercie. Madame la Ministre, tout ce que je vais vous dire, par rapport à ça quand on parle de déshumanisation. C'est bien parce que aujourd'hui les personnes qui se retrouvent devant un ordinateur ne sont pas forcément des jeunes et les plus anciens sont pas habitués. Ils préfèrent avoir quelqu'un parce que une fois qu'on est bloqué, soit un service informatique. Je vous prie trois que pour débloquer un dossier c'est très très difficile et ça il faut bien en tenir compte. Tout ce que je voulais vous dire, madame la Ministre, c'est que on a la délégation des collectivités territoriales qui fait à un boulot formidable et et ça il faut en tenir compte et c'est tout ce que je souhaite c'est que vous tenez compte de ses observations d'ailleurs qui a été fait côté effectué avec l'ensemble des collègues. Voilà, merci. Merci la parole est maintenant à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour huit minutes pour l'Union centriste. Monsieur le Président Madame la Ministre madame la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, mes chers collègues. Avant toute chose. Je souhaite remercier. La présidente très dynamique présidente de la délégation aux collectivités territoriales. D'avoir fait le choix d'organiser ce débat, il est donc question aujourd'hui de l'État, territorial, autrement dit la présence dans nos vallées sur nos littoraux ou dans nos villes d'administration dépendant directement du pouvoir central. Longtemps, ce centre de gravité institutionnel et politique fut exclusivement à Paris. Fruit d'une idéologie jacobine une organisation centralisatrice les normes devait s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Mais l'impératif d'adapter l'application des normes aux circonstances locales l'impératif surtout d'efficacité des politiques publiques ont généré plusieurs vagues de décentralisation à l'instar des lois de faire de 83 82. Mais aussi l'émergence d'une différenciation territoriale, la première avec la loi montagne de 1985. bosser à une nette à territoriale que je préfère aujourd'hui appelé la France des sous-, préfectures. Cette politique de décentralisation et déconcentration a montré son efficacité dans les territoires. Cette France des sous-, préfectures ne tire pas de mon point de vue un bilan totalement satisfaisant. Le dernier rapport de la délégation intitulé la recherche de l'État dans les territoires et sans appel. Pour compenser la baisse des moyens financiers et humains est largement perceptible. Notamment dans les territoires les moins dotés. Les effectifs physique des directions départementales interministérielles ont perdu 36% de leurs effectifs entre 2011 et 2020. Cet état de fait directement responsable d'un sentiment d'abandon. Souvent par les élus locaux et spécifiquement par les maires ruraux les normes s'accumulent au même rythme que les responsabilités alors que les interlocuteurs des services de l'État se raréfient et que les finances locales sont toujours plus comme ça a été rappelé par d'autres interlocuteurs intervenant cet après-midi. Quel est le résultat de cet effet ciseaux une disparition des services publics de proximité. Une lassitude des citoyens. Le rapport sur les services déconcentrés de l'État met également en valeur le manque de lisibilité institutionnel pour les élus locaux. à travers le questionnaire des rapporteurs. Il est indiqué que 64% des élus locaux considèrent que les agences de l'État sont trop nombreuses cette appréciation est partagée par les préfets et les sous-préfets dans une proportion encore plus conséquente, 80%. C'est bien connu, plus les effectifs diminuent plus les services se multiplient. Ainsi pour un maire d'une commune rurale, il est souvent complexe d'appréhender l'organisation territoriale de l'État. Encore la semaine dernière dans mon département lors de visites de communes, les maires ont indiqué et m'ont confirmé que pour eux l'unique interlocuteur connu accessible. Aussi efficace que possible demeure le sous-préfet d'arrondissement. Le 3ème enseignement majeur du rapport s'avère être le manque de concertation. Plus de 4 élus locaux sur 5 estime ne pas avoir été suffisamment associés aux différentes réformes des services déconcentrés de l'État je m'inscris évidemment dans cette tendance statistique en affirmant que ce ce ressenti est transposable sur un grand nombre de politiques publiques. C'est d'ailleurs une des problématiques dont se saisira la mission d'information sur l'avenir. Des communes et du maire en France qui en elles-mêmes et sa création montre et signifie quelque chose au grand public et et à la Cour de nos collègues maires élus locaux. Non j'ai l'honneur d'être un des vice-présidents. Pourtant les local est à la République ce que le coeur et au corps humain, c'est le 1er récepteur réceptacle. Des attentes citoyennes comme pendant les gilets jaunes ou durant la crise Covid. C'est également le dernier le garant du dernier maître des politiques publiques et je pense que la proposition de loi portée notamment dans nos collègues Valérie Létard et Jean-Baptiste Leblanc sur l'objectif Jeanne le démontrera si besoin était. Madame le Ministre et je le dis également au gouvernement fait confiance aux élus locaux. Alors comment faire de l'État, territoriale, une réalité. Cela passe évidemment par un renforcement du couple bien aimé des Français. Le couple mère préfets maires, préfets de département. Parce que j'ai entendu les déclarations de madame, la Première ministre devant l'Assemblée des départs des des communautés de France indiquant que pour elle il y avait un nouveau couple territoriale qui était le préfet. De département. Avec le préfet de région pardon avec les présidents d'intercommunalités les préfets de département, ceci ne nous paraît pas être une ligne satisfaisante pour enraciner la confiance dans les territoires. Et maintenir une commune et des mères actif. Du côté de l'État. Le principe de subsidiarité doit permettre au préfet d'avoir des pouvoirs accrus. La disposition votée dans le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur va par exemple dans le bon sens. Désormais en cas de crise. Il s'agit d'élargir le Champ l'autorité fonctionnelle des préfets. Aux services et établissements de Roland, pas de leur autorité en temps normal. L'idée proposée et ça a été rappelé tout à l'heure par Françoise Gatel de faire en sorte que le Premier Ministre soit l'autorité coordinatrice et l'autorité fonctionnelle. du préfet dans le département me paraît aller dans ce sens d'une meilleure coordination des services et d'une lisibilité des politiques de l'État central dans les territoires. Il faut aussi réarmer en terme de moyens, les services déconcentrés de l'État pour être au plus proche des territoires ce réarmement des services de l'État doit s'accompagner par une meilleure lisibilité des champs d'action des services déconcentrés. Face à la jungle administrative des collectivités notamment celles possédant des personnels en nombre limité. Les communes rurales doivent pouvoir trouver l'interlocuteur adapté à leurs besoins. Un autre rapport de la délégation forts prolixes en la matière porte portant sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires recommande de positionner le sous-préfet d'arrondissement comme l'interlocuteur de 1er niveau sur les questions d'ingénierie. Je tiens à souligner pour être équilibré dans mon propos en bon centriste que je suis, que la création de sous-préfet complémentaire dans les territoires est une bonne chose et permettra notamment dans les territoires doté de peu de services préfectoraux. D'abord un interlocuteur de plus grande efficacité en proximité. Je crois aussi pouvoir dire et et et et rappeler si besoin était, que la question de la dotation des préfectures n'est pas suffisante. Il y a eu un une vraie hémorragie. Du nombre de collaborateurs dans des services importants pour les maires et pour les collectivités locales que sont par exemple les DDT dont les effectifs ont fondu comme ont fondu comme neige ces dernières années. Or ce sont des interlocuteurs précieux du quotidien pour les politiques liées au droit du sol pour les questions de l'égalité pour les questions de contentieux ou de précontentieux pour les collectivités et les maires en particulier, je ne veux pas passer sous silence non plus. La situation des personnels des des défis. Comment voulez-vous que les collectivités puis gérer correctement avec des comptes public, avec des régies si elles n'ont pas la possibilité d'avoir des interlocuteurs de proximité en nombre suffisant. Et pas simplement regroupés dans le chef-Luc département. Des instances temporaires ont été aussi mis en place. Durant la crise sanitaire. Je pense en particulier à toute la concertation menée par les délégués des ARS sur les questions de santé. Durant cette période, je crois qu'il faut tirer enseignement de cette efficacité, et faire en sorte que les délégués d'ARS puissent être davantage soutenu et avec beaucoup plus d'autonomie dans les territoires. Je terminerai, madame la Ministre par 2 interpellations. La première, vous avez dit à plusieurs reprises l'importance de pouvoir effectivement travailler par la différenciation territoriale chiche sur la question de la compétence eau et assainissement. Allez-vous enfin pouvoir Madame. La Ministre convaincre et vous convaincre avec le gouvernement de laisser la liberté locale agir dans les territoires et faire en sorte que les collectivités puissent choisir librement leur manière de s'organiser dans les territoires avec cette compétence soit dans un cadre intercommunal soit dans un cadre communal et ne nous faites pas le coup comme le Ministre ce matin de dire que ce choix là est largement conditionnée par des questions de sécurité d'approvisionnement d'eau et de sécurité et d'hygiène, de l'eau. Je crois que c'est un mauvais argument. Dernière question concernant le MFS. Qui sont finalement des guichets mis en place par les collectivités locales comme sous-traitant de l'État. Je vous invite également à nous garantir que dans la durée les financements pour le financement de ses collaborateurs qui sont des collaborateurs des des des collectivités territoriales seront garantis dans la durée parce que recruter sur un statut ensuite ne plus avoir les financements. Je crois que ça peut être aussi un danger fort pour nous MFS demain et pour les collectivités locales qui en sont les responsables. Je vous remercie. Merci cher collègue. Et Madame la Ministre, vous avez 2 minutes pour. Répondre à notre collègue. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Arnaud, Les propos élogieux que vous avez tenus à l'égard des sous-préfets d'arrondissement rappeler qu'nous avons de des sous-préfets ruralité des sous-préfet France 2030 et nous avons là des serviteurs de l'État qui sont. En partenariat étroit avec nos élus locaux vous l'avez souligné vous avez souligné un certain nombre. D'actions que vous avez jugé efficace au 1er rang desquels vous l'avez pas dit mais je souhaite le souligner Petites Villes de demain qui est un programme de laine, c'était très efficace dans les sous-, préfectures, que vous avez cité et vous avez dit c'est pas totalement. On peut faire mieux. La réponse est oui, on peut toujours fait mieux, on va faire mieux, on doit faire mieux mais ensemble et donc c'est l'objet de ce débat dont personnellement je me félicite pour essayer de prendre toutes les idées. Que nous n'avons pas encore saisi et qui nous semblent pertinentes pour faire mieux au service de nos citoyens des élus locaux bien sûr mais des citoyens. Vous appelez de vos voeux que nous fassions confiance aux élus locaux. Un sénateur juste avant a rappelé une sénatrice là. L'engagement de Jean Castex. Je veux dire à quel point la Première ministre. Est elle aussi dans une véritable relation de confiance et à quel point pour elle le couple mère préfet est important même si elle a souligné à quel point le couple préfets présidents d'intercommunalités avait du sens comme vous le savez les compétences sont différentes. On était, on a vu l'efficacité du couple mère préfet sur des sujets sanitaires et ce couple mère-préfet il est très précieux dans plein de domaines qui sont du Champ de la compétence du maire sur des sujets qui sont compétence intercommunale très important de effectivement aussi tisser du lien entre le préfet, le président d'intercommunalités. Moi je ne pense pas en bon centriste que vous êtes qu'il faille les opposer. Ensuite je voulais souligner. En conclusion, parce que vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Le fonds vers le fond Vert il a cet immense merci. Vertu d'être au service. De nos territoires de nos élus locaux, d'être à la main des préfets et de servir des investissements au service de la transition écologique et de la transition énergétique. C'est un, un fonds qui est interministériel, il est extrêmement précieux très apprécié pour finir le financement de MFS merci madame total soutien pour faire en sorte que. Il soit un peu prolongé, merci. Merci monsieur Arnaud. Oui le ministre, je suis d'abord les gendarmes qui sont là parce qu'on a besoin aussi de force accident de départements les gendarmeries sont précieuses dans nos départements. Vous n'avez pas répondu mais j'en suis pas surpris sur la question de la compétence. Oh, ça tombe bien, nous avons une PPL peut être une deuxième peut être une troisième et puis nous allons organiser avec nos amis d'Arnaud avec Françoise Gatel avec de nombreux sénateurs très clairement on ne va pas vous lâcher sur le sujet parce que. L'eau effectivement, par définition ça passe rapidement mais je je pense aussi que l'eau est une façon de fructifier les territoires et de faire pousser de belles graines. Donc je pense que sur ce sujet-là, on ne lâchera rien et je regrette effectivement. Cette fuite en avant, si vous me permettez, toujours cette métaphore. Tout à fait. Liées à l'eau parce que ce sujet-là il viendra de toute façon on vous propose madame la Ministre, d'être à côté des locaux et de prouver par l'exemple, le fait que l'on peut laisser la liberté locale de choix à s'organiser dans le cadre de du territoire de la proximité. Prenez, prenez au rebond cette proposition généreuse constructive et puis nous vous applaudiront avec beaucoup beaucoup beaucoup d'efficacité et nous remercieront ce gouvernement nous avons entendu. Merci cher collègue. je vais donner la parole maintenant à au président Jean-Claude Requier pour cinq minutes pour le groupe RDSE. Monsieur le président m'la ministre madame la présidente de la délégation aux collectivités territoriales mais sa collègue j'ai déjà eu l'occasion de dire je vois c'était tribune dans une vie antérieure, j'ai été professeur d'histoire géographie. Mais le sujet retenu pour le débat de ce jour, l'État territorial ni réalité. Me rappelle les Bonnesoeur d'un terminal et les sujets du bac philo. Car vous le savez les historiens et géographes et les violences M. souvent s'écharper sur des concepts et sur des récits afin de déchiffrer des défricher ce qui relèverait du mythe ou du réel d'une illusion ou du vécu. Autant dire que l'intitulé du débat à tout pour me plaire

visitant la France en particulier, ou s'agit-il plus largement de modèles théoriques abstraits bien entendu je comprends l'esprit de la formule. Elle vise le rapport de l'État, territoire ou à ces territoires et plus spécifiquement. Le rapport les services déconcentrés de l'État et les collectivités, les Un moyen finalement de nous confronter à l'ambiguïté du lien entre le territoire de l'État et les territoires dans l'État. Bref, vaste programme que votre assemblée ne craignent pas l'affronter, je m'en réjouis par cette expression, nous poursuivons les travaux déjà engagés à 2016 par le Sénat. Suite au rapport d'information rendue par Éric Doligé et Marie-Françoise Pérol-Dumont. À l'époque, qui dressait le constat suivant. Les services déconcentrés de l'État sont confrontés à une succession de réformes qui remettent périodiquement en question leurs modalités d'réalisation leur prix action et leurs moyens matériels et humains plusieurs le profession métier ressorti parmi lesquels ceux de maintenir la proximité d'. Administration déconcentrée avec les collectivités territoriales, mais surtout de donner aux collectivités, les moyens de surmonter la complexité de l'organisation administrative et de ses procédures. Il y a quelques semaines. Nos collègues Agnès cavalier et Éric Kerrouche sont chargés de dresser un nouveau bilan sur ces questions via un nouveau rapport qui émane d'ailleurs toujours sur ce thème de l'État, territorial je souligner à qualité d'un travail aussi observé que notre assemblée qui assis dans son rang de chambre des territoires, mais surtout il en ressort que les problématiques dégager dès 2018 demeure pour l'essentiel les mêmes à ce jour. C'est tout particulièrement le cas de l'ingénierie une territoriale qui compte du de poser de nombreuses difficultés dans nos collectivités et en particulier dans les petites communes et communautés de communes de notre ruralité, symbole de la diversité territoriale de notre pays. Là-bas, les acteurs locaux élus agents font le constat régulier d'une baisse de compétences des services déconcentrés de l'État entre le groupe le groupe RDSE il est forcément sensible et nous avions souhaité apporter une réponse avec la création de la une, c'était en 2018. Celle-ci trouver son origine dans l'insuffisance. Voire l'absence des moyens d'engineering elle ainsi que le programme comme peut quitter les procédures accrues par la multiplicité des intervenants et des opérateurs.

l'manque encore de quoi nous occuper pour ces prochaines années afin de mettre en place des dispositifs qui favoriseront la bonne administration de nos territoires et cela naturellement venir de l'état aussi hein. Conclusion et pour revenir sur intitulé du débat, il faut choisir entre Mirage l'irréalité. Je dirais qu'une idée d'un État territorial dans au moins à représenter la réalité quand transformer. Et alors son cap, celui de l'administration homogène collaborative. Services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales à vouloir décrire. Et à s'expliquer cette notion d'État territorial nous découvrons enfin finalement un moyen d'analyser les sources du mal qui encore en compte nos administrations

Merci. Merci cher collègue. Et pendant que vous. Prenez votre place je passe la parole à Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la présidente. Monsieur le sénateur Riquier vous aborder. Plusieurs sujets le sujet. De l'administration déconcentrée auprès des collectivités territoriales, les difficultés d'ingénierie territoriale et vous appelez de vos voeux plus de simplifications sur les difficultés. et vous appelez de vos voeux sur le maintien de l'administration déconcentrée auprès des collectivités. Je veux redire ce que j'ai déjà dit et je dire à quel point le gouvernement renforce les moyens de l'État je vous avez dit que je lis seraient les cinq sous-préfecture qui ont rouvert leurs portes Château-Gontier en Mayenne Clamecy dans la Nièvre Montdidier dans la Somme Somme Rochechouart dans la Haute-Vienne et Nantua, dans l'Ain, plus une nouvelle sous-préfecture qui a été créée à Saint-Georges en en Guyane, ensuite je l'ai déjà dit mais je veux le redire après des années de diminution effectivement d'effectifs aucun emploi n'a été supprimé sur le périmètre de l'ATE l'administration territoriale de l'État en 2021 2022. Et la création de 350 ETP supplémentaires qui est prévu en 5 ans, dont 43 dès cette année, plus 30 postes de sous-préfet créer par redéploiement des postes de sous-préfet à la relance dans les départements ruraux plus la mise en place de sous-préfet référent thématique, je ne le répète pas plus la mise en place de 200 brigades de gendarmerie et je suis un peu triste que nos gendarmes sont partis mais en tout cas je voulais le saluer très amicalement la création de la haine. C'était, vous l'avez cité, c'est pour nous le lieu dans lequel s'incarne le choc d'ingénierie que nous voulons apporter. À nos collectivités territoriales, De vos voeux que ces moyens soient renforcées ces réalités, nous avons doublé nos effectifs et ça dès le 1er semestre 2023. Par les effectifs de délégués de proximité, ce sont ces représentants de la haine. C'était qui seront dans. Les préfectures nous en aurons a minima, un par région pour avoir un interlocuteur privilégié ingénierie pour toutes les collectivités locales y compris les plus petites, puisque je vous confirme que nous travaillons avec la haine. C'était sur un programme visant à servir les plus petites de nos communes françaises qui ont bien besoin d'ingénierie. C'est d'ici un mois que dans le cadre de France ruralité de ce nouveau souffle de l'agenda rural j'aurais plaisir à venir vous en parler si vous le souhaitez. Si madame la mini-je vous remercie,

quant au sous-préfecture. Je suis un serveur un fervent défenseur des sous-, préfectures, dans le monde rural parce que les maires retrouvent appui conseil auprès des sous-préfets et des sous-préfète.

Monsieur Riquier. Et maintenant la parole à notre collègue Agnès Canayer du groupe les républicains pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre madame la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, mes chers collègues si une réforme de l'État, territoriale et une décentralisation vont de Pair. Il n'y a pas de décentralisation réussie sans une déconcentration pertinente. C'est pourquoi je regrette la méthodologie défaillante des trop nombreuses réformes de l'État déconcentrer depuis 15 ans. La présidente Gatel a eu raison de rappeler l'enchaînement frénétique et l'empilement des réformes au point de donner le tournis aux élus locaux et de désorienter les agents de l'État eux-même si encore cette frénésie de réformes s'accompagner d'évaluation régulière et d'une analyse des retours d'expérience. On pourrait à la rigueur la suivre mais hélas ce qui est frappant dans ce mouvement perpétuel, c'est que la réforme suivante n'est jamais précédé d'une évaluation sérieuse, rigoureuse documentée de la réforme précédente. La mission d'information que nous avons menées. Avec mon collègue Éric Kerrouche a permis de souligner cette lacune. Elle met en évidence l'invoque distraction profonde des maires et des autres élus locaux. Alors que 61% des élus locaux considèrent que la réforme de l'organisation de l'État et souhaitables 82% regrette de ne pas avoir été associés à ces réformes qui les concernent pourtant en priorité. À cela il faut encore ajouter que plus de la moitié des maires notamment ceux représentant les communes de moins de 1000 habitants, estime que l'offre de l'État s'est dégradé où est défaillante dans leur territoire ce hiatus est d'autant plus préjudiciable que le véritable cours couples mère-préfet avait fait ses preuves tout particulièrement pendant la crise sanitaire sac hein chez ces pardon dans cet hémicycle le rôle essentiel des maires et de leur équipe dans la réponse efficace et de proximité. Aujourd'hui, les élus locaux. Nous ne sont plus dans la défiance envers l'État, territorial, au contraire, ils attendent de lui qu'il soit un véritable partenaire un accompagnateur plus attentifs. C'est pourquoi une clarification du rôle de l'État dans nos territoires est désormais indispensable. Il est urgent de mieux répartir les compétences de l'État sur la base de deux principes essentiels, la subsidiarité et la différenciation. C'est à cette condition que l'État pourra irriguer tout le raid territoire jusqu'au dernier kilomètre la contractualisation entre l'État et les collectivités représente une modalité intéressante et va dans le sens d'une souplesse recherchée. Elle permet de sortir de la logique des appels à projets trop technique pour les petites communes et qui impose un cadre strict bridant leurs initiatives. Au lieu de les soutenir rendent plus effectifs la relation mère préfet renvoie également au déminage de certains sujets de tension. Il est parti n'en est particulièrement vrai de celui des conditions d'attribution de la DETR, et de la de la dotation de soutien. À l'investissement local. Actuellement le préfet, le seul à décider du choix des projets pour les montants inférieurs à 100.000 euros alors que les élus n'ont pas toujours accès aux informations sur leurs dossiers déposés ni sur les attributions. Au terme de la mission d'information menée au nord de la délégation aux collectivités territoriales. Nous avons proposé. Davantage de transparence dans l'attribution des dotations. S'agissant de l'accompagnement des projets et des investissements locaux. La question du devenir de l'ingénierie territoriale se pose celle-ci a longtemps été la figure de proue de l'État dans les territoires. Chacun se souvient notamment du rôle des DDE toutefois. Depuis la disparition de l'assistance technique de l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, l'offre d'ingénierie de la part de l'état se trouve amoindrie pour ne pas dire déstabilisé. On peut même s'interroger sur la capacité de l'État, entretenir et à pérenniser son expertise technique. Il n'est pas anodin de constater comme un tiers d'ingénierie les communes les moins peuplées recours surtout au département, voire aux intercommunalités qui ont développé leur propre expertise. Parallèlement, les plus grandes collectivités se tournent davantage vers des prestataires privés de manière accessoire vers l'État et ses opérateurs. Certes la NTT marque un projet intéressant, mais il ressort de notre enquête, qu'elle souffre d'un vrai déficit de notoriété auprès des élus locaux. Par ailleurs, l'offre d'études qu'elle propose n'est souvent pas suivi des financements nécessaires pour mener à bien des projets, il faut y remédier. En conclusion et pour revenir au titre de notre débat. L'État territorial a longtemps été une réalité structurante pour ne pas en être réduit à devenir un mirage. Il doit être guidée par une vision claire et s'alimenter des recommandations de notre rapport j'espère Madame la Ministre que vous saurez vous en inspirer. Je vous remercie. Merci. Collègue et Madame la Ministre pour 2 minutes. Monsieur le président. Merci mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente, madame la sénatrice Canayer vous aborder plusieurs sujets la nécessité de proximité je ne renouvelle pas mes propos sur la façon dont le gouvernement renforce les moyens de l'État. Territorial comme vous l'avez intitulé je veux dire quelques mots complémentaires sur la une c'était qui a pour objectif d'instituer une logique de guichet unique au plus proche des territoires et si certaines critiques, notamment du fait de sa jeunesse. L'. A été ont été pointés par le l'excellent rapport du Sénat la haine c'était a connu aussi de nombreuses réussites notamment dans l'accompagnement des collectivités dans leur besoin d'ingénierie. Donc ces 1600 j'ai pas encore donné ces chiffres petite centralité de moins de 20.000 habitants, accompagné par le programme Petites Villes de demain et 906 postes de chef de projet subventionné. Sur votre droite, voilà. Pour Action coeur de ville, ces 5 milliards d'euros mobilisé sur 5 ans 234 communes sur 222 territoire métropolitain et ultramarin et 312 ORT signé au 15 octobre 2022 sur le sujet de l'évaluation, ça ça introduit mon 3ème point qui est la générique. J'ai déjà citée sur lequel je travaille depuis juillet, la Première ministre, comme vous le savez, m'a permis d'aller voir ce qui se passait réellement sur le terrain pour évaluer j'ai autant que vous mesdames et messieurs les sénateurs. L'intime conviction que nous devons encore plus évaluer l'efficacité de nos politiques publiques avant d'embrayer sur de nouvelles lois de nouveaux textes de nouveaux programmes, c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois c'est la Première ministre il me l'a demandé et c'est donc pour cela que va émerger quelque chose qui j'espère sera efficace mais on commencera à l'évaluer dès l'été 2023. Dès la fin 2023 pour voir comment réorienter si certaines actions n'étaient pas aussi efficace dans les ruralités que nous le souhaitons. Vous appelez de vos voeux. Plus de subsidiarité. Moi j'ai envie de vous dire, on peut toujours faire plus et mieux, je suis d'accord avec vous mais la fin des appels à projets. Le le le le fait que le Fonds Vert sur la main des préfets cette déconcentration telle que nous la voulons est telle que les préfets la mettre en oeuvre pour moi et tu un 1er fort signal et puis pour, pour ce qui est de la différenciation. Je veux vous dire à quel point aujourd'hui. Je suis fière et heureuse de porter un projet de loi ZRR. Version 2 acte de pour janvier 2024. Qui est vraiment une loi qui porte en son sein la différenciation de notes. Toi. Merci madame la ministre madame Canayer. Oui merci à la ministre sur la une, c'était effectivement on voit aujourd'hui que c'est un progrès mais qui a qui est largement perfectible mais en ce qui concerne l'ingénierie. C'est un peu à l'image de l'État aujourd'hui qui est dispersée dans ses réponses dispersés dans ses actions et je pense que un des enjeux forts pour donner de la lisibilité de la clarté et aide véritablement dans l'accompagnement des élus locaux. C'est d'une meilleure coordination de cette offre sur les territoires. Quant à l'évaluation. C'est vrai que c'est un sujet fort et récurrent. Il est important avant d'introduire toute nouvelle politique de ne pas reproduire ce qui s'est passé, à savoir l'addition et le mille-feuilles de réformes réformes sans aucune évaluation mais j'attire votre attention, madame la Ministre sur le fait que le baromètre ne peut en aucun cas être un outil d'évaluation, on ne peut pas évaluer uniquement par les chiffres, on ne peut pas évaluer uniquement par la quantité mais il faut une véritable évaluation qui porte sur la qualité de l'action qui est menée. Merci cher collègue. Et maintenant, la parole est à notre collègue Éric Kerrouche pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la présidente de la délégation Madame la Ministre, mes chers collègues, en entendant mon collègue de la majorité gouvernementale. Monsieur puis je me disais que ça doit être confortable de vivres dans le monde. De Oui-Oui territoriale. Pourtant. Madame la ministre. Il est tout à fait légitime de se poser la question de savoir si l'État a encore la moyen les moyens de ses ambitions dans nos territoires se poser. Se poser cette question est relativement étonnant pour un pays qui, depuis la loi du 28 pluvieux en huit a donné une place particulière à justement la place de l'État, territoriale et pourtant celui-ci cet été territoriale suscite des doutes des critiques. La mission de d'informations que nous avons pu conduire avec Madame Agnès Canayer pointe effectivement de, de nombreux enjeux. Et je me contenterai ici d'évoquer la question des moyens et de de l'organisation. Rares sont les champs de l'action publique qui ont connu autant de réformes que celui dont nous parlons. Mais cette spécificité trompeuse loin d'être un signe de vitalité et de bonne santé. Elle traduit surtout un malaise profond des objectifs qui n'ont pas été atteints d'où des remises en chantier répéter à un rythme qui s'accélère. À chaque fois la réforme de l'État, territoriale, et pourtant sous-tendu par une ambition louable clairement affiché, on veut améliorer le fonctionnement des services on vaut mieux répondre à la demande d'État dans les territoires. La réalité constatée et très différente puisque c'est celle d'une baisse continue des moyens de l'État. Les élus ne s'y trompe pas, d'ailleurs, 2 sur 3 estiment que le service public s'est dégradé sur leur territoire et près de 60% considèrent que les moyens des services déconcentrés sont insuffisants. Je vous rappelle également et c'est révélateur que 70% des membres du corps préfectoral, que nous avons interrogées estiment aussi que les moyens humains qui sont à leur disposition sont insuffisants. Il est d'ailleurs très difficile de reconstituer les chiffres des effectifs de l'État dans nos territoires, changement de périmètre suppressions de direction recréation rattachement à différents ministères tendent à brouiller les cartes il est impératif que le ministère de l'Intérieur se dote d'outils de suivi de l'ensemble des personnels déconcentrée. Qui lui ont été rattacher ces dernières années au travers notamment des directions départementales interministérielles. Malgré tout, on l'a déjà dit, les chiffres sont parlants, baisse de 15.000 fonctionnaires dans les DDI entre 2011 et 2012 ans entre 2011 et 2022, pardon, une baisse donc de 36%. La plupart du temps ces coupes sont censés avoir été compensé avec, dit-on, une organisation plus efficiente des gains de productivité. La diffusion de nouveaux outils technologiques. Pour autant, nous ne pouvons pas le savoir puisque il y a des suppositions. Mais rien n'est évalué ex Post. Contraire dans les auditions que nous avons mené les exemples de dégradation des services abonde. Cette politique dictée par une perspective qui est purement comptable montre les limites forte et je ne veux en prendre qu'un seul exemple celui du contrôle de légalité. On doit s'interroger sur la façon dont ce service est rendu aujourd'hui les préfectures, vous le savez de contrôle plus depuis bien longtemps l'ensemble des actes des collectivités locales et en fait. Utilise. Les actes à enjeu. Donc en gros la commande publique ces actes budgétaires et la gestion des ressources humaines. Or, même dans ce cadre, hé bien l'état d'atteintes pas ses objectifs qui frôle peut-être neuf sur 90% mais en tout cas pas l'intégralité de ce qui devrait être fait. Dans d'autres pays. Tout se passe comme si l'État territorial était resté figé dans une réalité qui ne correspond absolument plus à celle des collectivités locales. L'effet d'inertie est considérable dans certains départements, dans certaines régions, les effectifs des des services de l'État ne correspondent plus à la réalité du terrain mais un héritage du passé. Un récent rapport de la Cour des comptes. Ah, vous le savez conforter ce constat que nous avions déjà dressé dans notre rapport. Il faut sortir de ce carcan pour adapter l'État territoriale aux besoins contemporains. Vous avez parlé Madame la Ministre des sous-, préfectures qui ont été touchés de plein fouet par la RGPP. C'est très bien d'en réouvrir six sans c'est sans commune mesure avec les besoins qui serait nécessaire sur l'ensemble des territoires et dans chacune des sous-, préfectures, que. La carte des sous-, préfectures n'a pas été revue en profondeur, en tout cas depuis la réforme Poincaré de 1926 alors que depuis les périmètres, y compris ceux des collectivités territoriales ont été modifiés et qu'il conviendrait sans doute d'en tenir compte, tout en garantissant l'autonomie et les moyens de ses sous-préfecture. Je vous remercie. Monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente, monsieur le sénateur Kerrouche. Je vais épargner aux sénateurs présents. La poursuite de ce que j'ai appelé dans dans dans certains échanges parce que j'ai beaucoup apprécié ce débat. Mais ce que je pourrais appeler un dialogue de sourds. C'est-à-dire que moyens insuffisants. Difficile de compter. Qui sont les agents de l'État. Nous accuser de brouiller les cartes. Aucune évaluation or poste cette politique elle est comptable et cetera et cetera donc je vais pas vous redire tout ce que j'ai dit qu'ils vous laissent penser que mon intime conviction est totalement orthogonal, avec ce que vous avez dit ce que je simplement dire c'est que moi j'essaie de travailler. Avec des peut-être. Des gens que vous intitulez ou que vous appelez dès oui oui territoriale mais moi je j'ai beaucoup de mal à travailler avec des moins moins territoriale parce que le verre en France, il est tout le temps à moitié plein plein ou à moitié vide, tout le temps. s'il était toujours plein. Hé bien on aurait des citoyens heureux on aurait pas la France très clivée que nous avons aujourd'hui, on aurait pas des citoyens révoltés, on aurait pas des parlementaires révolté oui, rien n'est parfait. Cher monsieur, oui, tout peut être amélioré mon bureau vous êtes ouvert. Mais moi je préfère travailler avec des gens qui sont constructif pour essayer de faire évoluer les choses qu'avec des gens qui pointe tout ce qui va mal, même si dans ce qui va mal, il y a un certain nombre de choses qui sont tout à fait réalité qui doivent être améliorés. Je vous remercie.

Alors Madame la Ministre j'entends tout ce que vous dites mais je vais vous rappeler quelque chose de simple, il y a un sociologue qui s'appelle Émile Durkheim, qui a dit quelque chose qui est très important dans la méthode de de de sociologie en sciences sociales, c'est que les faits sont têtus. Et que les faits nous les avons pointés dans le rapport que nous avons rendu avec Madame Canayer. Vous pouvez les refuser sélectionner les critères qui a priori vous satisfont. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Et après, la question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord, pas d'accord. La question de. Elle est toute simple dans le ministres c'est quel niveau d'exigence. Nous avons vis-à-vis de l'État, territoriale et est-ce que nous avons envie que celui-ci soit à la hauteur du rôle qu'il devrait remplir dans les territoires. Vous dites que vous avez calmer les baisses d'effectifs depuis 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a eu un quinquennat avant donc la question c'est pas de dire que tout va mal Madame la Ministre mais c'est de voir la vérité en face et à partir de cette vérité d'essayer de tracer un chemin et avec tout le monde Madame la Ministre pas seulement avec ceux qui vous font plaisir politiquement. Merci monsieur Kerrouche. La parole est maintenant à notre collègue Mathieu Darnaud pour cinq minutes. Pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, chère Françoise Gatel. Il faut feindre que tout change pour que rien ne change. Madame la ministre, je me permettrai de prendre cette célèbre réplique du guépard car elle me semble aujourd'hui de circonstance en effet j'ai le sentiment, depuis que nous débattons ici même. De la constitution de la haine, c'était des maisons France service. De la déconcentration de l'État d'entendre à peu près toujours les mêmes intentions venant du gouvernement et pour couper court toute de suite. À une réplique que vous pourriez m'opposer me faire de ne pas être objectif. Permettez-moi de prendre quelques exemples concrets. Mado à ce que vient de dire mon collègue Éric Kerrouche. Les faits sont têtus. Vous parlez de la réussite des Maisons France service nous ne la contestons pas. Je m'empresse simplement de vous dire madame la ministre que les maisons de France services sont là pour remplacer des services de l'État qui ont disparu avec le temps notamment les trésoreries et beaucoup d'autres. Donc ce n'est pas une offre nouvelle, c'est une offre différente qui remplacent des services qui existait auparavant. Vous parlez du réarmement de l'État, territorial Madame la Ministre alors moi je vous invite très clairement puisque vous êtes encline à faire des déplacements et c'est très bien je le salue à venir dans mon beau département de l'Ardèche. Qui vous permettra de mesurer que les annonces faites par le gouvernement notamment au centre des impôts de on a parlé de la, des, des FIP où il avait été annoncé 50 moyens supplémentaires, nous attendons toujours le 1er de ses moyens. Je vous invite à venir dans la sous-, préfecture de L'Argentière ou de Tournon-sur-Rhône, pour voir que cet État territoriale dont vous parlez. Oui, il a besoin d'être armé mais réarmer avec des moyens humains et cela nous l'attendons de pied ferme. Vous évoquez aussi. Le fait de permettre aux zen, c'était de se rapprocher et de nourrir ce lien de proximité avec les élus, là encore, nous l'attendons, je rappelle qu'ici, nous avons toujours fait preuve du plus grand pragmatisme lorsqu'il s'est agi de débattent sur la haine c'était nous appelions de nos voeux qu'un état de l'ingénierie réelle sur les territoires soit opéré pardon de vous le dire, nous l'attendons toujours et nous attendons surtout que les actions qui soient mises en oeuvre sur notre territoire. Vous avez parlé de Petites Villes de demain. Puisse au delà des moyens d'ingénierie qu'elles généreront. Aussi et appelé de nouveaux moyens financiers car l'ingénierie. C'est bien, faut-il encore que l'état puisse donner des moyens complémentaires pour permettre la réalisation de ce qui sera produit par par l'ingénierie. Enfin et c'est peut-être là. Le noeud essentiel du problème, le noeud gordien. On ne peut pas parler d'état territoriale. Si on ne donne pas aux préfets et aux préfets de département les moyens de coordonner l'action de l'État. Et alors, vous me permettrez Madame le Ministre très clairement d'opposer. De choses à ce que vous venez de de dire tout d'abord, vous nous dites. Et là je suis prêt puisque vous nous y invités à venir débattre avec vous approfondir le sujet. Parler du du pouvoir dérogatoire des préfets alors pardon je le cherche. On a été avec Madame Gatel, rapporteur du texte, le pouvoir dérogatoire du préfet Madame la Ministre il il. Pour qu'il puisse voir le jour. Faudrait-il encore avoir une réforme constitutionnelle et notamment une réforme de l'article 72. Vous dites que finalement, le préfet a pu coordonner l'action de l'État pendant la crise. Ah bah moi je prends à témoin les 35.000 maires de France qui ont dû lire avec attention les protocoles scolaires sanitaires pour ouvrir ou fermer les écoles et vous verrez combien les préfets ont eu comme difficultés à agir pour pouvoir justement interpellé et intervenir vis-à-vis des services de l'éducation nationale. Tout ça c'est une réalité, une réalité vécue, une réalité qui va parler au maire alors. Vous nous invitez à être pragmatique, chiche. Soyons pragmatiques et être pragmatique c'est aussi demandé au gouvernement de mettre en application ce qu'il nous promet Ayant rappelé que nous avons été avec Françoise Gatel, rapporteur du texte 3DS que n'avons-nous pas entendu de la part du gouvernement d'engagements pris pour permettre déconcentration pour permettre ce réarmement il se renforcement des pouvoirs de coordination de coordination des préfets, les seuls sujets qui ont vu le jour. On était de donner une suite pratique et législatives aux propositions que le Sénat a fait l'Office français de la biodiversité et faire du préfet, le délégué de l'Office français il y a bien dire c'est c'est ici que ça a été décidé vouloir mettre en place un pouvoir dérogatoire. Nous l'attendions malheureusement nous l'attendons encore. Donc ce sont des choses très claires, très pragmatique. Nous sommes prêts à avancer mais puisque aujourd'hui le débat nous invite à répondre. Pour savoir si l'État territorial est une réalité ou un mirage. Moi je suis un défenseur de l'État, territoriale, je pense que c'est effectivement une réalité. Qu'en revanche vos engagements sont souvent des Mirage. Je vous remercie.

qui a changé de place. Est revenu à la sienne. Il s'était rapproché mesdames et messieurs les sénateurs, donc. Tout d'abord je vais venir en Ardèche. Entre les mois de mars et avril mai fin avril au plus tard, je serai venue chez vous. Première réponse positive. Réarmer les. Nos territoires. J'ai simplement envie de dire. Poursuivre ce que nous faisons ne ne ne ne pointons pas nos différences. Je pense que les chiffre que je vous ai donné sont très objectif. Vous les jugé insuffisant. On va y travailler, on est tous convaincus que les services de l'État en régions peuvent être renforcée pour travailler toujours et encore avec les élus locaux localement là où je veux juste souligner un point mais je pense que vous l'avez en tête, mais quand vous dites l'ingénierie. C'est bien que j'ai un peu rappeler tout ce que nous faisons les les l'argent qui a été injectée qui continue d'être injecté avec les améliorations qu'on va porter Allen cette sur la recommandation du Sénat et que je vous ai parlé du programme en ingénierie dans les petits villages. Je pense que je, je vous ai rassuré sur le fait qu'en ingénierie. On va poursuivre et s'améliorer. Par contre vous dites le lien avec l'investissement, bon je veux bien que vous me parlez de 1024 il y aura le temps pour y travailler mais 2023. DETR et décide de milliards d'euros structurellement chaque année la DETR a doublé ces 10 dernières années et le Fonds Vert c'est juste 2 milliards de plus ça double encore donc c'est 4 milliards d'euros qui vont être injectés. Certes les 2 milliards de fonds Vert avec une très forte composante écologique transition écologique et transition énergétique mais c'est quand même 4 milliards d'euros pour faire suite à quoi ben aux travaux d'ingénierie que les maires vont conduire avec le soutien de la haine, c'était que nous finançons en en en très grande partie donc su pour conclure juste et pour pas dépasser mes deux minutes sur le pouvoir dérogatoire. J'entends que que vous dites parce qu'aujourd'hui j'ai demandé le chiffres c'est 350 fois que les préfets ont fait appel à ce pouvoir dérogatoire qu'ils ont. Vous dites, c'est insuffisant. Moi je vous avoue que je suis incapable de vous dire si il faudrait qu'il déroge plus moins sur les sujets éducatifs sur lequel je suis totalement solidaire de ce que vous dites, il faut pouvoir adapter. Les politiques publiques que nous conduisons nationalement et que mon collègue pape poursuit d'ailleurs je le rencontre demain matin. Mais ce pouvoir dérogatoire. Il est là, on peut effectivement appeler de nouveau qui soit un tout. Bertrand

comme le mien avec le le désengagement progressif des des agences de l'eau. Je veux surtout concentré mon propos sur la question des préfets. Et et vous inviter comme vous l'avez fait notamment à l'occasion de l'examen de la loi 3DS ah vous inspirer les travaux du Sénat et notamment à l'excellent rapport. De nos collègues Kerrouche et canaille et je le dis parce qu'il correspond à une réalité. Il est le reflet des attentes de l'État, territorial, sur le territoire, mais plus encore des élus locaux qui attendent beaucoup de vous qui attendent surtout du congrès je vous remercie. Monsieur d'Arnaud. Donc maintenant nous nous nous acheminons vers la conclusion de de ce débat, donc je vais donner d'abord la parole à Madame la Ministre pour cinq minutes pour la conclusion générale. Puis ensuite à la présidente Françoise Gatel. Donc Madame la Ministre. les sénateurs. Voilà, vous pouvez le faire là si vous voulez, c'est la conclusion générale. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Mes premiers mots seront pour remercier. Françoise Gatel, la très dynamique, comme cela a été dit, présidente de la délégation aux collectivités territoriales c'est un vrai plaisir. Tu es un véritable aiguillon. Aiguillon constructif. La délégation qui t'accompagnent aussi vous dire que c'est. Pour moi. Avec beaucoup de sincérité que je vous remercie d'avoir mis ce sujet État territorial entre mirage et réalité. À l'ordre du jour de ce jeudi 9 février. Je veux aussi dire à quel point com Jean-Claude Requier. Il y est à quel point je me suis intéressé à l'esprit de la formule et ce titre est était. Intéressant. Les débats peuvent toujours être encore plus approfondies encore plus nourris encore plus. Ambitieux, mais en tout cas pour moi c'est la première fois je conduis cet exercice et je dois vous avouer que je les conduis avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de notes.

Je vis ça comme un honneur d'avoir été invité à ce débat organisé à la demande de de la présidente Gatel et de la délégation. Alors vous connaissez mon attachement, vous ne le connaissais pas mais je vous le confirme aux collectivités territoriales à la ruralité aux élus locaux à l'initiative territoriale mais aussi au débat parlementaire. Ce débat, j'espère que nous pourrons le renouveler à de nombreuses occasions dans les semaines et mois à venir, convaincu que c'est ainsi que nous trouverons les solutions les plus adaptées aux difficultés que rencontrent nos concitoyens ce débat était aussi pour moi l'occasion de rappeler certains points de l'action du gouvernement à destination des collectivités territoriales, auxquelles je suis tout particulièrement Ce débat était aussi pour moi de rappeler à quel point le travail qui est fait par les préfets, les sous-préfets les services de l'État en régions sont efficaces. Notre pays a raison du contexte en raison du contexte international est confronté à une inflation importante qui touchent directement les collectivités notamment dans leurs coûts de fonctionnement. Les mesures que nous avons prises dans le PLF 2023 vise à réduire ces difficultés. La prolongation du bouclier tarifaire qui limite l'augmentation des coûts de l'énergie à 15% dans les petites communes. La mise en place d'un amortisseur électrique grâce auquel l'État prend en charge 50% des surcoûts de d'un prix de référence de 325 MWh la reconduction d'un filet de sécurité étendu à toutes les collectivités ou encore l'augmentation de la DGF de 320 millions d'euros pour la première fois depuis 13 ans, sont autant de mesures qu'il était urgent et indispensable de prendre pour moi c'est peut être ici même que résident les fondations de l'État, territorial dans sa capacité à accompagner chaque collectivité à ne laisser au con mais aucun maire sur le bord de la route en période de crise. Cette présence bienveillante. Doit être renforcée. Toujours plus et se mettre toujours plus aussi au service des collectivités territoriales qui sont elles-mêmes au service du bien commun et de nos concitoyens la volonté du président de la République et du gouvernement a été clairement affirmé et réaffirmé la réouverture de 5 sous-préfecture, je l'ai dit, la création d'une nouvelle sous-préfecture le déploiement de 2538 Maison de France service sur tout le territoire ou encore les mesures présente dans la Lopmi la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur avec le déploiement de plus de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires dans les territoires ruraux et périurbains démontre notre volonté de réimplanter l'État dans nos territoires, la création de la haine s'était créée il y a maintenant 3 ans marqué aussi cette volonté forte du gouvernement précédent, de rapprocher les moyens de l'État, des collectivités territoriales et même si j'ai pris connaissance avec attention du rapport du Sénat que vous m'avez remis hier et qu'il ne faut pas nier qu'il existe de véritables axes d'amélioration pour cette jeune administration son existence même va dans le bon sens. C'est pour cette raison que la haine c'était verra ses moyens en ingénierie doubler dans les territoires. Dès 2024, le marché de l'ingénierie sera par ailleurs déconcentrer afin de rapprocher le processus décisionnel des territoires et des et et les élus, comme vous le voyez la une c'était évolue grandit et se rapproche des territoires pour conclure je rajouterai que l'État n'oublie pas le volet investissement pour les collectivités territoriales, notamment avec le Fonds Vert. Ces 2 milliards d'euros supplémentaires qui seront à la main des préfets Vous l'aurez compris, la réalité de l'État, territorial, c'est un État qui accompagnent qui soutient qui aide les collectivités territoriales au quotidien ne voyait pas dans mes propos un élan d'auto-satisfaction. J'ai conscience des leviers qui restent à mobiliser mais je voulais aussi souligner ce qui avait été fait et bien fait aussi je mesure le chemin qu'il nous reste à parcourir ensemble les difficultés que rencontrent nos collectivités. Les défis qui se présentent à nous, ce n'est qu'ensemble que nous arriverons à progresser. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Et maintenant, pour conclure le débat. La parole est à la présidente Françoise Gatel. Monsieur le président. Merci mes, mes chers collègues, je veux vraiment remercier tous les collègues qui étaient présents aujourd'hui toutes les questions été extrêmement pertinentes et je profite aussi pour adresser mes remerciements à tous les membres de la délégation président requis. Moi j'ai aimé. Votre votre volonté de définir ce qu'est un débat et de définir le le sujet. Madame la Ministre. Alors je vous le dis avec beaucoup de d'amabilité et de gentillesse même la franchissent habituelle. Un débat est un espace de discussion pour construire sur un sujet, trouver des solutions alors que ça n'est pas un grand Oral. Et ça n'est pas non plus, on va dire un espace de justification, c'est-à-dire il n'est pas dans notre idée de faire un procès. Du gouvernement. Nous, notre souhait c'est simplement que la France, elle marche et que les maires qui portent de grandes responsabilités, puissent être accompagnées par l'État et alors à certains moments Madame la Ministre ça va peut-être pas vous plaire mais je vous le dis gentiment. Certains ont dit que c'est un après-midi d'oui oui moi je dirais pas ça, mais on était, ça me faisait penser les plus jeunes ne connaissent pas mais à ces séquences ou Elkabbach interrogeait monsieur Marchais et quel Abachidzé. Ce n'était pas ma question Monsieur marcher elle disait c'était ma réponse, bon moi je pense. Madame la ministre et vous l'avez dit, que le rapport qui a été fait par nos collègues Chamaillé et qui rouge il va à l'essentiel, c'est un travail de fond et qu'il doit être considéré comme une contribution positive et rigoureuse. À la réflexion, que le gouvernement même ce que je ne doute pas de votre intention et qui anime le président de la République puis sur nous faire oeuvre utile et être dans ces séquences en perspective de solution et je sais que c'est votre état d'esprit mais cet après-midi je le sentais pas trop. Alors ensuite, moi je pense qu'il y a et ça a été dit une exigence d'évaluation. Il faut évaluer ce que l'on fait et il faut encourager les expérimentations et je rejoins Agnès Canayer quand elle dit qu'un comptage ou un baromètre ne sont pas une évaluation. Est-ce qu'on peut avoir des évaluations qualitatives et Madame la Ministre, vous avez entendu ce que nous avons dit au départ, c'est que l'évaluation qui a été fait où la mesure de la satisfaction, ça n'est pas que celle des élus, c'est aussi celle du corps préfectoral qui est constitué de gens absolument remarquable. Alors je vous invite, madame la Ministre a participé aux États de généraux de la simplification nous nous organisons le Sesmat où nous voulons travailler ensemble avec des engagements clairs, y compris celui du gouvernement sur une fabrique de la loi qui soit efficace et efficient différenciation Madame la Ministre vous y croyez moi aussi j'y crois. Alors il y a le pouvoir réglementaire locale du préfet. OK. Et je vais reprendre ça gâche tout le monde mais c'est pas grave, c'est quand même un sujet l'eau et l'assainissement. Enfin si si on est encore en train de parler de ça c'est qu'il y a des problèmes et que l'eau et l'assainissement. Non, enfin l'eau n'a jamais coulé dans un périmètre administratif et nous ne disons pas que les communes doivent rester. Mais permettant de travailler à des solutions efficaces et que les autres Hautes-Alpes ne sont pas là la Bretagne enfin madame la mini-, je redis ce que n'ait pas, répondit à cet excellent de recommandation du rattachement du préfet. Au Premier Ministre parce que ça permettrait d'avoir une unité. De la voix de l'État. Une chaîne de commandement, on peut appeler ça un chef d'orchestre dont on a vu l'efficacité pendant. La crise sanitaire. Madame, je ne serai pas plus long, moi je suis heureuse de ce temps que nous avons eu. peut-on Madame la Ministre et je vous fais pas de griefs personnel je sais votre volonté d'écouter de comprends mais que l'on comprenne que compte les sénateurs expriment des choses c'est pas juste pour embêter le monde où passer un après-midi récréatif. C'est vraiment parce que nous avons des convictions. Nous voulons des solutions et que nous vous proposons, vous l'avez dit, madame la ministre, de faire ensemble. Alors si nous pouvons avoir un prochain débat vraiment qu'il soit un débat et non pas. Un jeu de ping-pong, je serais heureux et ravi. Merci Madame la Ministre merci mes chers collègues. Mes chers collègues, je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu le mardi 14 février à 9h 30 pour les questions orales. La séance est levée.

Merci